La séance est reprise. Madame la ministre, mes chers collègues, avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote.

Vous êtes heureux de l'apprendre, mes chers collègues : je vous l'annonce ! Derrière un projet de loi qui, comme son nom l'indique, se doit d'aborder en premier lieu le financement des comptes sociaux transparaît l'adoption de mesures concrètes et nécessaires pour l'avenir de notre pays et de son système social.

trouvent les tenants, dont je suis, d'une hausse de la CSG. Cette mesure nous paraît plus juste ; en particulier, elle garantit une solidarité intergénérationnelle, raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité exonérer les retraites au-delà d'un certain seuil.

hausse. Alors que notre système de protection sociale est fondé sur la solidarité intergénérationnelle, l'article 7 de ce texte avait selon moi trouvé un équilibre.

mais aussi toute une génération qui a voulu vivre au-dessus de ses moyens. Venons-en maintenant à la branche maladie. Les mesures concernant l'innovation ont fait consensus. L'innovation en matière organisationnelle- téléconsultation et télé-expertise -entre dans le droit commun grâce à l'article 36. innove aussi en matière de rémunération, en sortant du « tout paiement à l'acte » au profit de rémunérations forfaitisées ou de l'intéressement collectif au niveau des établissements. Tout cela reste guidé par la recherche d'une meilleure pertinence des actes.

prévention du cancer du col de l'utérus est elle aussi encouragée ; je vous avais interrogée la semaine dernière sur le sujet. Enfin, on lutte contre le tabagisme par une fiscalité dissuasive. Concernant la branche famille, le Gouvernement a décidé de donner la priorité aux familles les plus pauvres, en particulier monoparentales.

les faire évoluer vers un système plus social. De cette réflexion découlera un vrai choix de société en matière de politique familiale. À propos de la branche vieillesse et du secteur médico-social, là encore, il nous faudra aborder la question à l'aune de l'allongement de l'espérance de vie.

il reste à mes yeux un texte de transition, en attendant les grandes réformes qui feront débat : la retraite, l'autonomie et, de façon plus générale, le vieillissement. On ne fera pas non plus l'économie d'une réflexion sur les allocations familiales, je le répète. Le principal point d'achoppement sera le financement. Demain, nous nous retrouverons en commission mixte paritaire, afin de discuter de la façon dont chacun souhaite construire ce budget.

Au-delà de l'aspect purement financier, c'est aussi une affaire d'éthique que d'inscrire notre système de protection sociale dans la durée. En reprenant la dialectique de Max Weber, j'opposerai à une éthique de la conviction, certes respectable, une éthique de la responsabilité.

amplifie les choix antérieurs, dont on a pourtant pu constater les effets désastreux, de la loi HPST à la loi Touraine. Durant cette semaine, ce sont en réalité deux visions de l'avenir de notre système de sécurité sociale qui se sont affrontées, deux projets de société diamétralement opposés. La vision, que vous avez présentée, madame la ministre, avec « tact et mesure », pour plagier les termes de l'article du code de la santé publique censé lutter contre les dépassements d'honoraires- dispositions notoirement insuffisantes à transformer la sécurité sociale en un système étatique et fiscalisé qui prendrait en charge uniquement les prestations sociales des plus précaires : les familles monoparentales, les privés d'emploi, ou encore les retraités les plus fragiles.

Ce projet de privatisation de la santé rejoint totalement celui de la droite. Notre vision est aux antipodes de ces choix : nous défendons un système de protection sociale pour toutes et tous. Certes, il doit évoluer, mais il faut continuer à le faire reposer sur ses principes fondateurs : la solidarité, l'universalité des prestations, la gestion démocratique et le financement par la cotisation sociale.

fixé à 2,3 % pour 2018, et jusqu'en 2020, soit un manque à gagner de 4 milliards d'euros par an, vous m'ave z répondu : « Le système dysfonctionne, non par manque d'argent, mais parce que nous n'avons pas fait les réformes nécessaires. Je souhaite un changement de philosophie. Je vous propose une réforme de fond qui réduira la gabegie et concentrera les dépenses sur les soins utiles. »

qui travaillent au quotidien à l'hôpital avec des moyens en baisse ; ils jugeront ! Malgré votre refus de voir la réalité en face, madame la ministre, ils vous diront qu'ils subissent le non-remplacement des départs à la retraite et les fermetures des services. Ainsi, au CHU Henri-Mondor de Créteil, Créteil, de lourdes menaces pèsent sur les services de chirurgie cardiaque et hépatique, six ans après une lutte emblématique qui avait permis de sauver le premier. Ces personnels soignants, toutes catégories confondues, sont en souffrance,

Vous dites qu'il faut réduire la « gabegie » quand ces agents parlent de « pénurie ». Là encore, ils apprécieront vos propos ! Refuser obstinément d'aller chercher des recettes nouvelles, notamment en mettant un terme aux exonérations de cotisations patronales et en taxant la finance, c'est ne pas créer les conditions pour désengorger les urgences, ne pas desserrer l'étau asphyxiant les hôpitaux, ne pas revitaliser et améliorer la psychiatrie de secteur, ne pas lutter contre les renoncements aux soins, ne pas combattre les déserts médicaux, ne pas garantir le suivi des personnes en perte d'autonomie, ne pas assurer un maillage territorial

Vous menez une politique des « deux poids, deux mesures ». Aucun article de ce PLFSS n'est consacré aux moyens de combattre la fraude patronale, qui s'élève pourtant à 20 milliards d'euros, tandis que vous traquez la fraude sociale sans commune mesure. Le Défenseur des droits a d'ailleurs mis en garde sur ce qui serait des erreurs de déclaration, plus que des volontés intentionnelles de fraude. Tandis que vous justifiez la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les 100 foyers les plus riches, soit une perte de 3,4 milliards d'euros pour satisfaire les biens communs, vous vous acharnez sur les salariés et les retraités, en augmentant la de 1,7 %. Nos amendements, conjugués à d'autres, ont permis de limiter un peu cette injustice. Ainsi, la Haute Assemblée, bien qu'elle n'ait hélas pas voté sa suppression, a tout de même rejeté la hausse de la CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité, pour les personnes dédommagées au titre de la prestation de compensation du handicap et pour les artistes auteurs. Malheureusement, ces avancées, ainsi que les reculs que nous avons évités sur les articles portant sur la politique familiale risquent d'être balayés à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, comment ne pas regretter que la généralisation du tiers payant soit remise à plus tard ou que vous n'ayez pas entendu, madame la ministre, les nombreux Français qui auraient préféré un débat plus approfondi sur les conditions de l'extension vaccinale avant d'être mis devant le fait accompli Enfin, nous serons très vigilants, dans les mois à venir, sur les engagements que vous avez pris concernant la limitation des prix des médicaments. Mes chers collègues,

comme nous l'avons démontré avec mon collègue Dominique Watrin tout au long de ces débats. Toutefois, ni le gouvernement Philippe-Macron ni la droite sénatoriale- on l'entend avec le brouhaha qui règne dans l'hémicycle -n'en ont la volonté politique. Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera

madame la ministre, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, après les débats le plus souvent constructifs

le groupe Union Centriste du Sénat a reçu votre projet de loi avec un positif. En effet, nous nous retrouvons en grande partie dans la vision de la politique sociale que vous comptez mener tout au long de ce quinquennat. Nous soutenons l'impératif d'équilibre des comptes sociaux, avec un ONDAM maîtrisé et, surtout, les objectifs et la méthode pour y parvenir. Ceux-ci tiennent en quelques mots : pertinence des actes, prévention et innovation.

L'approbation que nous apportons à votre politique générale trouve néanmoins ses limites avec l'article 7. Le Sénat dans sa grande majorité et notre groupe en particulier se sont opposés à la taxe additionnelle à la CSG pour les pensions des retraités supérieures au SMIC. En effet, si nous souscrivons à la politique et à la philosophie générale de l'article consistant à redonner du pouvoir d'achat aux actifs, sa mise en oeuvre apparaît très complexe et la participation des retraités ne nous semble pas opportune. En tout cas, elle est plutôt perçue comme injuste par les retraités eux-mêmes. Plusieurs solutions de substitution ont été envisagées. Le groupe centriste avait notamment proposé de la remplacer par une légère hausse de la TVA, ce qui aurait permis de faire contribuer les consommateurs étrangers au financement de notre système de protection sociale. Pour ma part, je regrette que l'on ait laissé passer l'occasion de faire converger le taux normal de CSG applicable aux actifs et aux retraités pour un même niveau de revenus, en exonérant les pensions de la taxe additionnelle. Au-delà de cette question, madame la ministre, il faut poursuivre la réflexion sur la diversification des sources de financement de la sécurité sociale, car nous ne pourrons pas éternellement augmenter la CSG ou baisser les cotisations sociales. Nous avons également supprimé, sur l'initiative de notre collègue rapporteur Élisabeth Doineau, l'article 26 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE. Par la suppression de cette mesure, qui ne revêtait aucun caractère d'urgence, nous avons souhaité en appeler à une réflexion d'ensemble sur la politique familiale de notre pays. Le principe d'universalité a été remis en cause par votre prédécesseur, madame la ministre. Vous avez souhaité engager une réflexion sur la politique familiale : nous en attendons les fruits avec impatience. Nous avons supprimé deux mesures, certes parmi les plus emblématiques, de votre PLFSS, mais nous regrettons aussi les votes négatifs du Sénat survenus, contre l'avis des rapporteurs et de la commission, sur certaines dispositions des articles 7 et 8. Nous avons soutenu l'article 8 et, à cet article, les mesures de transformation du CICE en diminution des charges sociales en faveur des entreprises. pourront ainsi renouer durablement avec la compétitivité. Nous vous avons également soutenue, madame la ministre, dans votre projet de supprimer le régime social des indépendants, le RSI, qui avait perdu la confiance des assurés depuis ses débuts, il faut le dire, chaotiques. le Gouvernement n'a pas le droit à l'erreur et nous vous remercions d'avoir accepté plusieurs amendements pour garantir un portage politique fort en la matière et un pilotage efficace pour que cette réforme offre de offre de meilleures conditions de recouvrement, notamment aux assurés. Enfin, je voudrais de nouveau affirmer notre soutien sur trois axes de votre projet de loi : la prévention, l'encouragement l'encouragement des innovations et la pertinence des actes. La prévention est essentielle, car elle permet d'éviter de nombreuses pathologies chroniques et, parfois, des épidémies. C'est ainsi que nous avons soutenu l'obligation de vaccination. Nous vous invitons surtout à renforcer la médecine scolaire, qui est dans une situation alarmante. L'innovation est au coeur de votre politique en matière d'organisation des soins, avec la promotion de la télémédecine, par exemple, ou pour lutter contre les déserts médicaux. Pour éviter les 30 % d'actes inutiles ou redondants que vous dénoncez, il faut espérer que cette année verra la mise en oeuvre du DMP, permettant aux acteurs de terrain de proposer les soins les plus pertinents et les plus économiques. Madame la ministre, mes chers collègues, la situation des finances sociales de notre pays s'améliore,

Le Gouvernement ouvre de nombreux chantiers : stratégie nationale de santé, lutte contre les déserts médicaux, politique familiale et réforme systémique des retraites- celle-ci devra rassurer les 40 % des Français qui craignent de ne pas percevoir à l'avenir de retraite. de retraite. Notre groupe sera un partenaire exigeant. Nous vous soutiendrons de manière constructive, si la concertation avec le Parlement s'affirme encore plus.

mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, quel regard le groupe socialiste et républicain porte-t-il sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, à l'issue d'une semaine de débats où des visions bien différentes de l'avenir de notre protection sociale se sont dessinées ? Un regard contrasté, mêlant satisfaction, déception et interrogation. satisfaits quand le Sénat supprime la hausse de 1,7 point de la CSG applicable aux retraités- nous avions déposé un amendement identique à celui qui quand les personnes dédommagées au titre de la prestation de compensation du handicap sont exonérées et qu'une compensation de cette hausse de CSG est mise en place pour les artistes auteurs.

Dans la troisième partie du projet de loi, relative aux recettes, nous nous félicitons de décisions obtenues, soit avec notre appui, soit sur notre initiative. Je citerai fin de l'inégalité de traitement devant les charges sociales des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, pour les tâches effectuées au domicile de personnes âgées ou en situation de handicap possibilité de rendre cumulable le dispositif d'année blanche avec le dispositif d'exonérations partielles applicables aux jeunes agriculteurs l'offre « service emploi association » accessible aux entreprises de moins de 20 salariés ; l'exonération de la taxe sur les véhicules de société pour les véhicules fonctionnant au superéthanol E85

aux dépenses : la suppression de la baisse de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, qui avait été envisagée par alignement du montant et des plafonds de ressources de l'allocation de base sur ceux du complément familial réforme de la tarification de la dialyse, très attendue par les personnes concernées, à travers un forfait unique, adapté au profil de chaque patient, dispositif qui permettra le développement de la dialyse à domicile suppression du dispositif d'ajustement à la baisse, au-delà d'un plafond de dépenses, des prix et tarifs des dispositifs médicaux et des prestations associées ; le rejet d'un amendement de la majorité sénatoriale visant à supprimer le pécule constitué par le cumul des allocations de rentrée scolaire des enfants confiés aux services d'aide sociale à l'enfance. quatre motifs de déception et de vive opposition à travers des rejets d'amendements. Tout d'abord, le tiers payant généralisé, devenu généralisable. C'était, madame la ministre, un signe fort adressé aux familles ayant des revenus modestes, un instrument facilitant l'accès aux soins, déjà en place dans de nombreux pays européens. Nous serons attentifs au suivi du rapport qui sera remis en mars prochain.

1 janvier, l'abaissement de 30 % à 20 % du taux des cotisations patronales sur la distribution d'actions gratuites par les grandes entreprises. Nous confirmons, madame la ministre, notre soutien à l'ensemble des mesures de prévention.

consultation gratuite de prévention du cancer pour les femmes âgées de 25 ans et l'obligation vaccinale portée à 11 vaccins, que nous approuvons. Nous confirmons Nous confirmons aussi notre appui attentif aux mesures d'expérimentations organisationnelles et à l'inscription de la téléconsultation et de la télé-expertise dans le champ ordinaire de l'assurance maladie. Enfin, le caractère universel de notre protection sociale, confirmé en 2016 avec la protection universelle maladie, est accentué par la disparition du RSI.

modes de rémunération, liens avec la ville, organisation des urgences et financement des investissements. un risque de déstabilisation de notre système des ATU, qui est pourtant envié dans le monde entier, car il permet un accès rapide des malades aux médicaments en innovation de rupture.

notre jugement ouvert sur les propositions formulées nous conduira à nous abstenir sur le vote final de ce projet de loi. Ce projet de loi de financement n'est pas un acte isolé. Il doit être lu en miroir avec d'autres décisions ou positionnements. J'ai en tête, d'un côté, les déclarations radicales du président de Goldman Sachs,

la pauvreté. Entre le libéralisme ultime, qui ignore la dimension humaine, et un pays refermé sur lui-même, nous croyons fortement qu'il existe un espace politique pour affronter les réalités d'un monde global, en gardant les fondations de solidarité, de justice sociale et de lutte contre les inégalités. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, notre assemblée se réunit aujourd'hui pour donner un avis final sur l'ensemble du PLFSS pour 2018, au travers duquel sont proposées la maîtrise des dépenses de sécurité sociale, la mise en place d'innovations et d'expérimentations pour la résorption des déserts médicaux, enfin l'anticipation des transformations techniques numériques de la santé. Notre groupe soutient les objectifs de renforcement de l'accompagnement des plus fragiles et de retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale en 2020 et de la CADES en 2024. Le Gouvernement envisage un effort de limitation de l'augmentation des dépenses de sécurité sociale à 2,1 % pour l'année prochaine, avec une diminution du déficit global d'euros en 2017. C'est une première étape sur la route d'un équilibre des comptes en 2020, et vous avez, madame la ministre, notre entier soutien dans cette démarche. L'article 7 porte sur l'allégement- 3,5 points -des cotisations sociales des salariés

sur les pensions de retraite à 1,2 point. Cette mesure avait un coût- 1,3 milliard d'euros -, mais nous est apparue comme un entre-deux raisonnable, un juste équilibre entre l'effort demandé par le Gouvernement et l'amendement tendant à abroger cette hausse de CSG sur les pensions de retraite, avec une

l'exclusion de la hausse de la CSG pour les personnes qui perçoivent la PCH et la suppression du remplacement du taux de cotisation maladie des exploitants agricoles par un taux progressif en fonction du revenu. L'article 8, relatif au soutien aux entreprises, taxe sur les salaires, le CITS, en un allégement pérenne des charges patronales, dans la limite de 2,6 SMIC. Nous avons soutenu la proposition d'autoriser les EPCI à bénéficier de l'exonération des charges sociales en contrepartie du travail au domicile des personnes âgées et handicapées. Nous avons aussi soutenu les exonérations des cotisations sociales des vendangeurs. Nous avons voté en faveur de la fusion de la

pour une protection collective. Je rappelle la gravité de la coqueluche chez le nouveau-né : dix morts ont

avec la nouvelle fiscalité sur les boissons sucrées. Quant à la politique familiale, nous avons été sensibles à la proposition faite à l'article 25 de majorer le complément du mode de garde de 30 % pour les familles monoparentales et nous avons voté, par la suite,

mesures portant sur la branche médico-sociale- personnes âgées et personnes handicapées -, dont le quatrième plan autisme. Notre groupe a étudié avec intérêt les propositions d'expérimentations pour l'innovation de notre système de santé. Nous fondons beaucoup d'espoirs sur l'article 35,

coconstruction avec les acteurs de terrain, consultations avancées en maison de santé, médecins spécialistes et médecins partagés, téléconsultation. Comme vous, madame la ministre, nous ne souhaitons pas de coercition pour les jeunes médecins. Mais l'État doit avoir un objectif : un médecin à plein-temps ou à temps partiel dans chaque maison de santé. C'est un enjeu de santé publique

Nous avons voté en faveur de la dernière partie du texte, relative aux nouvelles dépenses de sécurité sociale pour 2018. Néanmoins, la suppression pure et simple de la hausse de la CSG sur les pensions de retraite, représentant peut entraîner des difficultés quant à l'équilibre du PLFSS et du PLF. Notre groupe proposait une solution intermédiaire pour éviter cette impasse financière et nous espérons que la commission mixte paritaire permettra de conclure un accord équilibré maîtrise des dépenses publiques et le souci de moduler la charge des retraités dans le cadre de leur participation à l'effort de redressement des comptes publics. Monsieur le président, madame la ministre,

je suis heureux de pouvoir porter la position du groupe du RDSE sur ce PLFSS pour 2018, le premier de ce nouveau quinquennat. Avant toute chose, le groupe du RDSE tient à saluer la qualité et la richesse de nos débats, avec une mention toute particulière pour vous, madame la ministre. Vous avez pris le soin de répondre de manière argumentée à chacune et à chacun d'entre nous, avec la volonté, bien entendu, de convaincre et une sincérité certaine. Nous remercions également les différents rapporteurs de notre commission des affaires sociales. pour en venir à l'essentiel, s'agissant de l'augmentation de la CSG pour les retraités, la très grande majorité du RDSE n'est pas convaincue qu'un retraité dont le revenu mensuel net atteint 1 394 euros puisse être rangé dans la catégorie des retraités aisés ... C'est la raison pour laquelle le Sénat a adopté plusieurs amendements, dont celui du RDSE, visant à supprimer Si cette mesure devait être rétablie, il nous semblerait opportun de relever le plafond des ressources à environ 1 600 euros par mois. De même, la mise en place d'un taux progressif pour la cotisation maladie des exploitants agricoles nous semble inappropriée et c'est en ce sens que nous avons produit un amendement visant à supprimer Je rappelle que le taux de 3,04 % était un engagement pris par l'État en 2016. En métropole comme dans les outre-mer, la profession est en pleine crise, et ce taux progressif n'aurait fait qu'amplifier davantage le sentiment de détresse. Avant le second examen du texte à l'Assemblée nationale et la probable réintroduction de ces deux mesures, le RDSE, si vous le permettez, madame la ministre, vous invite à bien prendre en considération les échanges qui ont animé notre hémicycle ces derniers jours et qui nous avaient conduits à supprimer ces dispositions. Sur l'initiative de notre commission des affaires sociales, un article additionnel après l'article 11 a été inséré dans le texte, instaurant des mesures exceptionnelles pour les entreprises de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, mon territoire. Il s'agit de mesures légitimes qui vont permettre aux entreprises locales, actuellement en souffrance, de respirer et de relancer l'activité économique au plus vite. C'est essentiel pour nos deux territoires. Je veux prendre le temps de remercier le Gouvernement d'avoir respecté ses engagements vis-à-vis de ces deux territoires sinistrés et la commission des affaires sociales d'avoir bien voulu porter cet amendement, absent du texte transmis par l'Assemblée nationale. Au sujet des vaccins, le RDSE a apprécié tout particulièrement la réponse que vous avez faite à notre collègue Véronique Guillotin lorsqu'elle vous a interrogée au sujet du papillomavirus. nous serons vigilants, madame la ministre, quant au respect de l'engagement que vous avez pris dans cet hémicycle de saisir la Haute Autorité de santé et de travailler avec Santé publique France pour relancer des campagnes de vaccination. pour 2018, madame la ministre, mes chers collègues, a également subi des transformations à l'Assemblée nationale. Je voudrais revenir sur une disposition, fruit d'un amendement du rapporteur général : l'article 13 créant la contribution sur les boissons sucrées. Même si nous souscrivons à l'objectif de ce dispositif tendant à renforcer la lutte contre l'obésité et la surconsommation de produits sucrés, nous considérons qu'il comporte malheureusement un certain nombre de limites si l'on peut contrôler le taux de sucre dans des boissons sucrées, par exemple, comment s'y prendre pour les pâtisseries et les autres produits ? Et des cas où le sucre est présent en faible quantité dans des produits, alors qu'il ne devrait pas s'y trouver, comme dans la vinaigrette industrielle ? Nous voyons dans cette mesure un énième recours à la fiscalité comportementale, qui regroupe entre autres la hausse des prix du tabac, encore présente dans ce texte, la multiplication des radars ou encore la taxation des véhicules polluants. Ce type de fiscalité à deux inconvénients majeurs, à notre sens : il n'impacte quasiment que les populations les plus défavorisées, puisque les populations les plus aisées ne seront pas gênées par la hausse des prix ou des taxes il ne va pas favoriser une meilleure consommation, puisque les plus défavorisés vont se reporter en grand nombre sur des produits de substitution ou sur le marché noir. Taxer, d'accord, mais ne devrions-nous pas prioritairement axer nos efforts sur l'éducation ? L'éducation, madame la ministre, touche équitablement chacun, quel que soit le milieu social ou le niveau de rémunération. Comme de nombreux collègues, nous avons été déçus de voir la réforme du tiers payant, qui aurait bénéficié aux plus nécessiteux et aux plus vulnérables, supprimée avant son entrée en application. Si nous comprenons les problèmes de faisabilité que vous avez soulevés, nous restons convaincus que la suppression pure et simple n'était pas la seule solution possible. Nous verrons avec le recul. Avant d'en venir aux éléments absents de ce texte que nous aurions aimé voir abordés, nous voulons saluer l'adoption de plusieurs mesures pleines de bon sens la réflexion sur un organisme financier dédié à l'investissement immobilier des établissements de santé publics ; l'accès aux dossiers électroniques partagés pour les pharmaciens biologistes la possibilité d'une tarification pour les dialysés en fonction du patient et non de la prise en charge. J'en viens maintenant aux mesures qui doivent réformer en profondeur notre système de santé

Nous espérons que le Gouvernement se penchera assez rapidement sur ces problèmes, dont nous n'ignorons pas la complexité. Nous aurons la possibilité d'en débattre dès le projet de loi de financement de la débat, parce que nous voulons aussi que notre pays avance, le RDSE, dans sa grande majorité, votera le texte amendé par notre Haute Assemblée.

le rapporteur général. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au nom de mon groupe, permettez-moi d'abord de saluer le travail du rapporteur général, Jean-Marie Vanlerenberghe, ainsi que de l'ensemble des rapporteurs, Catherine Deroche,

Les débats ont confirmé nos points de désaccord, notamment sur la hausse de la CSG, qui entraînera une baisse du pouvoir d'achat pour de nombreux Français. Nous avons fait le choix, en toute responsabilité, de supprimer cette augmentation lorsqu'elle n'était pas compensée.

nous considérons que le Gouvernement choisit la mauvaise voie : s'attaquer aux 8 millions de retraités, que vous considérez comme des nantis, c'est mettre à mal la solidarité intergénérationnelle. Je ne reviendrai pas sur toutes les mesures, plus catégorielles, qui ont été adoptées par le Sénat portant sur des baisses ou des allégements de charges. Mais si ces débats ont eu lieu, madame la ministre, c'est bien la preuve que vos réformes ne sont pas abouties.

Nous avons exprimé des motifs d'inquiétude sur les conditions de rattachement des indépendants au régime général et nous avons essayé d'apporter quelques réponses. Tout d'abord, cette réforme ne doit pas se traduire, pour les travailleurs indépendants, par plus de complexité. Or le passage d'un interlocuteur unique à trois interlocuteurs n'est pas synonyme de simplification. Cela a conduit le Sénat à prévoir des guichets dédiés à l'accueil et à l'accompagnement des indépendants. Quant au niveau des cotisations, nous avons souligné que les travailleurs indépendants, qui attendaient de cette réforme une baisse des charges, vont être déçus : à prestations égales, l'adossement au régime général conduira, au pis, à une augmentation des charges, au mieux, au, comme l'affirme le Gouvernement. Pour notre groupe, la suppression du RSI doit s'accompagner, à court terme, d'une simplification à la fois de l'assiette des cotisations, mais aussi des modalités de leur recouvrement. Nous resterons donc vigilants quant à la mise en oeuvre de cette réforme. Nous avons également dénoncé la continuité avec les années précédentes en matière de politique familiale. L'an dernier, nous avions combattu la modulation des allocations familiales, qui signe la fin de leur universalité, et la réforme du congé parental. Ces deux mesures, qui représentent, à notre sens, des économies injustes au détriment des familles, n'ont malheureusement pas été remises en cause. Pis, vous poursuivez la casse de notre politique familiale avec la nouvelle baisse de la prestation d'accueil du jeune enfant, Notre politique familiale comporte, de longue date, de nombreux dispositifs destinés à répondre spécifiquement aux situations des familles dont les ressources sont les plus modestes. Il n'en demeure pas moins qu'elle accordait aussi à chaque foyer, indépendamment de son niveau de revenus, une forme de compensation des charges familiales. depuis le dernier quinquennat, cet élément constitutif fort de notre politique familiale est désormais dangereusement fragilisé- c'est le moins qu'on puisse dire. Notre désaccord s'est traduit par le rejet de la nouvelle baisse de la PAJE, qui nous semble injustifiée et inopportune au moment où le Gouvernement souhaite ouvrir un débat « apaisé » sur l'avenir de notre politique familiale. S'agissant de la branche vieillesse, notre collègue rapporteur René-Paul Savary l'a qualifiée dans son rapport de deuxième « homme malade » de la sécurité sociale. Nous avions contesté, l'an dernier, l'idée selon laquelle le problème des retraites aurait été réglé. Le retour à la réalité ne s'est pas fait attendre, sans pour autant que le Gouvernement en tire de conséquence. Nous souscrivons à l'objectif d'unification des cotisations et des droits, mais il s'agit d'un objectif de moyen terme, laissant entière la question de l'accentuation à très court terme des déséquilibres. Il faudra donc y répondre rapidement par une réforme paramétrique, sans attendre la mise en place d'une réforme systémique, d'autant que l'exercice sera nécessairement complexe à mener. de l'assurance maladie, madame la ministre, nous avons soutenu les mesures de santé publique et de prévention que vous avez proposées sur le tabac, la vaccination, les consultations de prévention pour les jeunes femmes. La suppression de l'obligation générale du tiers payant témoigne d'un changement d'approche indispensable vis-à-vis des professionnels de santé. Nous approuvons les mesures en faveur des nouvelles formes de prise en charge des patients, mais elles seront sans doute insuffisantes pour donner corps à cette ambition que nous partageons avec vous, madame la ministre, à savoir préserver l'accès à des soins de qualité sur notre territoire en rendant efficaces les modes d'organisation. Limiter l'intervention de l'administration à une juste régulation, redynamiser l'exercice libéral de la médecine, donner une plus grande autonomie de gestion aux hôpitaux publics, favoriser le travail complémentaire du secteur public et du secteur privé et réaffirmer le rôle de l'assurance maladie dans le financement de notre système de protection sociale sont autant de mesures illustrant le changement de cap que nous appelons de nos voeux. Ce changement de cap, nous ne le retrouvons que partiellement dans votre projet de loi. Nous n'avons pas pu illustrer ces mesures par des amendements, mais nous sommes convaincus que des mesures structurelles sont nécessaires. Permettez-moi de revenir quelques instants sur l'idée de donner plus d'autonomie de gestion aux hôpitaux publics. Le dialogue social mené aujourd'hui dans les hôpitaux souffre à la fois d'un excès de formalisme et d'un manque d'autonomie, ce qui ne permet pas d'adapter des décisions prises au niveau national à l'échelle locale ou d'innover. Cette innovation est cependant indispensable pour l'hôpital dans de nombreux domaines. Tout d'abord, en matière d'innovation technologique : je pense à la télémédecine, à la robotique, mais aussi à la médecine prédictive grâce au progrès de la génétique, qui contribuera à un parcours du patient plus personnalisé. Ensuite, en matière d'innovation organisationnelle : l'innovation technologique va, en effet, faire de l'hôpital un lieu de passage gérant les flux de patients. la mutualisation des équipements et l'approche collaborative doivent s'inscrivent dans cette nouvelle logique. Enfin, pour garantir la pérennité du système, il est nécessaire de repenser l'hôpital en dépassant les prés carrés, l'individualisme et la dispersion génératrice de coûts. Il faut au contraire développer une vision collaborative et compétitive de l'hôpital, autour de plateaux techniques communs et partagés par différents intervenants en la matière- publics, privés, chercheurs, industriels, etc. Nous sommes satisfaits de l'adoption de plusieurs mesures dont les bénéfices seront pour les patients. En matière de lutte contre les déserts médicaux, nous avons exonéré partiellement de cotisations vieillesse les médecins acceptant de reprendre ou de continuer une activité, afin qu'ils puissent cumuler activité libérale et retraite. En matière de dispositifs médicaux à domicile, nous avons supprimé le plafonnement du nombre de prestations fournies aux patients à domicile, qui aurait pour conséquence de les priver de ces de ces prestations et de freiner le développement de l'ambulatoire. Pour conclure, madame la ministre, mes chers collègues, nous restons très préoccupés par la situation des comptes sociaux. Nous avons tous le même objectif : l'égalité de toutes les Françaises et de tous les Français devant l'accès aux soins. Mais, devant l'ampleur des réponses à apporter,

Madame la ministre, mes chers collègues, il va être procédé, dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement, au scrutin public solennel

je proclamerai le résultat. La séance est suspendue.

de très grande qualité. J'ai souhaité et j'ai pu chaque fois exposer mes convictions- essayer de convaincre, comme l'ont dit certains -, parfois avec succès d'ailleurs, puisque nombre d'amendements ont été retirés par différents groupes quand j'ai pu

J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale à la prospective a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

L'ordre du jour appelle le débat sur l'avenir de l'Institut français, organisé à la demande de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes très chers collègues, « il suffit de passer un peu de temps à l'extérieur de notre territoire pour le constater : toutes les puissances renforcent aujourd'hui les moyens de leur politique étrangère. Si nous voulons rester maîtres de notre destin et assurer notre souveraineté, il faut que nous disposions d'un instrument diplomatique efficace, agile et capable de défendre nos intérêts Monsieur le secrétaire d'État, sans doute ces phrases ne vous sont-elles pas étrangères : ce sont celles de M. le ministre Le Drian lui-même, prononcées il y a à peine quelques jours devant l'Assemblée nationale. J'y souscris pleinement. j'ai malgré tout le regret de vous dire que, en matière de diplomatie culturelle, nous avons depuis de trop nombreuses années été bercées de bonnes paroles, alors que, sur le terrain, nos outils se paupérisaient d'année en année et que, paradoxalement, le besoin et la demande de France n'avaient jamais été aussi importants-

À l'occasion de chacun de nos déplacements à l'étranger, nous ne manquons pas de visiter l'Institut français, l'Alliance française, le lycée français ou l'antenne de Campus France qui portent nos couleurs et nos valeurs dans le monde. Et nous suivons bien sûr avec attention l'offre audiovisuelle extérieure, qui fait partie intégrante de notre diplomatie culturelle globale. Tous ces opérateurs qui agissent sur le terrain, parfois dans des conditions difficiles, sont remarquables et je tiens à leur rendre hommage pour leur inaltérable engagement à valoriser la culture et la langue françaises, mais aussi à susciter les échanges et les coopérations interculturelles. d'État, que notre commission a créé, sur mon initiative, une mission d'information sur la francophonie au XXI siècle, qui a publié en début d'année un rapport sous la signature de nos collègues Louis Duvernois et Claudine Lepage. J'espère que ces travaux pourront utilement contribuer aux réflexions en cours dans le cadre du « Plan de promotion de la langue française dans le monde » récemment annoncé par le Président de la République. Revenons, mes chers collègues, au sujet qui nous réunit ce soir : l'un des fers de lance de notre diplomatie culturelle, l'Institut français. Le Sénat garde un oeil très attentif sur l'Institut, à la création duquel il a contribué en 2010. Vous savez que notre ambition initiale- j'ai une pensée pour Jacques Legendre -était de lui rattacher le réseau des instituts français, mais ce projet a fait long feu et son abandon nous laisse un goût d'inachevé. Plus grave, depuis sa création, chaque année sans exception, les moyens alloués à l'Institut français se sont réduits comme peau de chagrin. Est-ce ainsi que les gouvernements successifs ont entendu donner son envol au nouvel opérateur ? En 2018, certes, les moyens se stabilisent enfin, mais à quel maigre étiage ! Rendons-nous à l'évidence : l'Institut est aujourd'hui exsangue et ne peut plus assurer l'ensemble des missions qui lui sont confiées, en dépit de l'engagement exemplaire de ses personnels.

Depuis sa création, en 2011, l'Institut a vu son budget fondre de 24 %, ce qui, compte tenu de ses charges fixes, a conduit à diminuer ses crédits d'intervention de 35 %. Les coupes sont extrêmement alarmantes : 43 % de baisse au cours du précédent quinquennat pour le département du cinéma, cinéma, 44 % pour le département de la langue française, du livre et des savoirs, et même 55 % a pour le département de la coopération artistique ! S'agissant des collaborations de l'Institut avec les collectivités territoriales que nous représentons, les moyens alloués ont baissé de 35 % en à peine trois En février dernier, lorsque le contrat d'objectifs et de moyens de l'Institut français nous avait été soumis ici au Sénat, notre commission de la culture, de l'éducation et de la communication avait émis les plus grandes réserves : d'un côté, des ambitions immenses, auxquelles nous ne pouvions que souscrire ; de l'autre, s'agissant des moyens, des subventions notoirement insuffisantes sans aucune visibilité pluriannuelle, pour un opérateur qui porte pourtant la voix de la France et de la francophonie, qui valorise nos industries culturelles et créatives, qui promeut le français à l'étranger et qui, faute d'une rebudgétisation rapide, devra probablement baisser pavillon.

m'a paru utile pour évoquer ensemble les missions, les moyens et les perspectives d'avenir de l'Institut, mais aussi, car il ne faut pas les oublier, des alliances françaises, qui concourent également au rayonnement de la langue et de la culture françaises, avec des moyens toujours plus réduits. La question d'une nouvelle articulation entre l'Institut français et la Fondation Alliance française devra également être évoquée, mais prenons garde de nous précipiter sur des solutions simplistes dans le seul but de gérer la Mes chers collègues, je vous invite donc à un large débat pour que, collectivement, nous prenions enfin nos responsabilités et réfléchissions à bâtir une politique culturelle extérieure digne du grand pays qui est le nôtre. La parole est à M.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je partage entièrement les inquiétudes de Mme la présidente Catherine Morin-Desailly sur la trajectoire budgétaire de l'Institut français. Sachez que nous sommes, sur toutes les travées de cet hémicycle, collectivement inquiets de ce décalage grandissant entre les bonnes intentions, la bonne volonté des gouvernements successifs, et le manque criant de moyens. Nous avons besoin, monsieur le secrétaire d'État, non plus de bonnes paroles, mais d'actes, d'actes « sonnants et trébuchants », si vous voyez ce que je veux dire Je n'ignore pas la contrainte budgétaire qui est la vôtre- c'est aussi la nôtre ! Je suis, moi aussi, partisan d'économies courageuses sur le train de vie de l'État, mais taillons dans les dépenses de fonctionnement, et non d'investissement. je considère que la politique culturelle extérieure est un investissement, qui rapporte ensuite à notre économie culturelle, créative, touristique, mais aussi, tout simplement, industrielle. Bien souvent, et vous le savez aussi bien que moi, les succès culturels de la France à l'étranger précèdent et préparent ses succès commerciaux. Pour contourner cette contrainte budgétaire, il faudrait faire preuve d'imagination et développer, ici ou là, des solutions innovantes qui permettront à la culture française de garder sa place dans le monde. Ne pourrait-on, par exemple, envisager des regroupements, des mutualisations, à une échelle soit européenne, soit francophone ? Les actions conjointes franco-allemandes me semblent, à cet égard, particulièrement intéressantes. Je me suis laissé dire que, à Rangoon, l'Institut français de Birmanie partageait ses locaux avec le Goethe-Institut ... Mais peut-être pourrait-on aller plus loin qu'une simple colocation ? Le conseil des ministres franco-allemand de juillet dernier a d'ailleurs évoqué la création d'instituts culturels franco-allemands intégrés dans le monde, peut-être au Ghana, en Mongolie, en Tanzanie Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'État, nous en dire un peu plus et préciser quelle pourrait être le rôle de l'Institut français dans ces nouveaux dispositifs ? La piste d'une coopération renforcée avec des équivalents francophones me semble également à étudier

un rapport sur la francophonie qui formulait de nombreuses et intéressantes propositions pour une francophonie du XXI siècle. L'une de ces propositions était de « mutualiser nos actions, voire nos implantations culturelles et linguistiques, avec d'autres pays francophones En avril 2015, avec la commission de la culture, j'ai eu l'occasion de visiter la Maison Denise Masson à Marrakech. Cet établissement est le fruit d'une coopération non pas seulement franco-marocaine, mais Francophonie-Maroc. Ce qui est bon pour la francophonie l'est aussi pour la France, et je suis persuadé qu'il existe, avec nos partenaires francophones, de belles occasions à saisir pour continuer à faire rayonner la culture et la langue françaises de par le monde. Une telle proposition ne pourrait-elle pas s'intégrer dans le plan pour la promotion de la langue française dans le monde annoncé par le Président de la République le 2 octobre dernier ? La parole est à M.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce débat sur l'avenir de l'Institut français touche à une question fondamentale,

tous les continents. Mais cet héritage n'est pas immuable. Il doit être non seulement préservé, mais aussi transformé, modernisé et adapté aux réalités du XXI siècle. En effet, la concurrence est forte, démultipliée par la mondialisation de l'information et le tournant des réseaux sociaux. Elle nécessite que nous soyons très présents, sur tous les fronts,

Je ne reviendrai pas sur la trajectoire budgétaire évoquée par la présidente Catherine Morin-Desailly, mais la question des moyens est évidemment essentielle. Depuis sa création en 2011, l'Institut français a su imposer sa marque, comme symbole du rayonnement culturel de la France. Il est connu et remarqué dans le monde entier. Il faut d'ailleurs en remercier ses équipes et présidents successifs, qui ont su l'implanter dans le paysage culturel non seulement français, mais aussi mondial. mais aussi mondial. Au-delà de la seule culture française, l'Institut français encourage les échanges culturels à travers le monde, et se place ainsi comme un acteur important d'une diplomatie culturelle globale.

j'évoquerai quelques pistes qui seront autant de questions. Tout d'abord, la demande de culture française à l'étranger est multiforme et probablement variable selon les régions du monde, les pays et les publics, français ou étrangers. Y a-t-il toujours concordance entre l'offre de culture française à l'étranger et la demande exprimée ? Sans se limiter à cette approche, adopter une démarche empirique, fondée en premier lieu sur le terrain et les retours d'expérience, me paraît essentiel. Ensuite, pour une diffusion auprès de publics les plus larges possible, ne faut-il pas réfléchir aux synergies entre l'Institut français et les autres acteurs français à l'international ? Les opérateurs de l'audiovisuel extérieur- TV5 Monde, France Médias Monde -sont des partenaires naturels de l'Institut français. Quel est le nombre de collaborations entre l'Institut français et les opérateurs audiovisuels ? Peut-on évaluer leur impact en termes d'audience ? Cela doit être possible, même si c'est difficile. Peut-on encore augmenter ces partenariats afin de permettre aux opérateurs audiovisuels de bénéficier de l'expertise de l'Institut français, et accroître l'impact de notre politique d'influence ? Enfin, même si on ne peut évidemment pas réduire la diplomatie culturelle à cette dimension, elle est aussi un instrument de la diplomatie économique. Mes chers collègues, sachez que les exportations des industries culturelles et créatives françaises représentent 32 milliards d'euros. Comment l'Institut français est-il associé à cette dimension, qui est inséparable de son action ?

et la Fondation Alliance française. Ces deux structures sont dans des situations très différentes, puisque l'Institut français est un établissement public chargé de la mise en oeuvre de l'action culturelle extérieure de la France à l'international, parallèlement avec le réseau culturel de nos ambassades. La Fondation Alliance française anime quant à elle un réseau de 813 alliances locales, associations de droit local, qui réalisent plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et s'autofinancent à 96 %.

en train de mettre en place des offres numériques concurrentes, ce qui n'est acceptable ni financièrement ni politiquement. Il faut donc faire le contraire et développer la complémentarité de l'approche par la langue qui est celle de l'Alliance et de l'approche par la culture qui est celle de l'Institut français, puisque, on le sait, apprendre le français amène souvent à s'intéresser à la culture française ; réciproquement, s'intéresser à la culture française conduit souvent à apprendre le français.

ne doit pas être seulement un moyen de gérer la pénurie de ressources publiques ; il doit s'accompagner de moyens supplémentaires pour donner à la France le rayonnement culturel qui doit être le sien en raison de son histoire et de sa culture. La parole

Nous sommes réunis autour d'un sujet majeur, celui de l'influence, du rayonnement de notre langue et de notre culture, auquel, vous le savez, le Président de la République attache un un soin particulier : il a eu l'occasion de s'exprimer lors de la Conférence des ambassadeurs le 29 août dernier, en annonçant son souhait de mettre en place un plan ambitieux de promotion de la langue française, de défense du plurilinguisme. effet, nous sommes dans un monde ouvert et la langue française est elle-même ouverte, véritable passerelle vers autant de cultures qui en sont des affluents. Dans le contexte de l'élaboration de ce plan, toutes vos réflexions sont précieuses.

qui constitue un réseau très dense- vous êtes, en tant que sénateurs et sénatrices, souvent amenés à rencontrer les diplomates, les conseillers culturels et le monde associatif travaillant avec ce réseau

Nous travaillons aussi avec le Goethe-Institut dans le cadre du Fonds culturel franco-allemand, qui encourage des initiatives de coopération culturelle en pays tiers,

sur la coopération avec nos amis francophones. Renseignements pris, puisque vous avez évoqué ce sujet, je me suis tourné vers nos amis du Quai d'Orsay pour

complexe, mérite à tout le moins un sens diplomatique aigu. C'est pourquoi l'ambassadeur de France

Message reçu, mesdames, messieurs les sénateurs ! Vous avez émis le souhait d'une diplomatie culturelle ambitieuse qui permette à la France de jouer un rôle important dans ce monde multipolaire, où elle a une voix différente

Ses missions sont parfaitement complémentaires avec celles de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ainsi, comment le Gouvernement compte-t-il mettre à profit cette coopération, tout en assurant le maintien et le développement de ces deux structures ? La parole

180 suppressions de postes confirmées et 160 autres potentielles dans les écoles françaises, consécutives, entre autres, à l'annulation de 33 millions d'euros de

est consacré à un programme d'excellence qui semble se développer. Nous ne sommes pas contre ces programmes d'excellence, mais nous craignons une politique trop axée sur un certain élitisme.

débattre de l'Institut français, c'est évoquer la place de la culture française dans le monde. Dans une société en pleine mutation, le « modèle français », reconnu au fil des siècles, doit se réinventer afin de perpétuer le rayonnement de la France et de la francophonie. L'Institut français y contribue en exerçant une mission de promotion de l'action culturelle extérieure de la France en matière d'échanges artistiques, de diffusion dans le monde du livre, du cinéma, de la langue française, des savoirs et des idées. En 1906, lorsque Julien Luchaire a fondé le premier culturel français en Italie, à Florence, le jeune professeur de langues de l'université de Grenoble ambitionnait de créer « une maison, ouverte à la fois aux jeunes Français et à leurs pareils italiens, où ils travailleraient ensemble, se connaîtraient, nourriraient entre eux des liens qui s'étendraient aux familles, à la société de la ville ». En 2017, à l'heure où l'Europe est soumise à des tensions, cette connaissance commune est plus que nécessaire pour resserrer les liens des Européens. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires est particulièrement sensible à cette entreprise de coopération culturelle à l'étranger. Nous entendons donc y apporter une attention particulière à l'occasion de l'examen prochain du projet de loi de finances pour 2018. La question des moyens financiers de l'Institut culturel est l'objet de ma présente interrogation. Ainsi, monsieur le secrétaire d'État, j'ai constaté avec satisfaction que vous étiez conscient des difficultés financières rencontrées par les instituts dans le monde et que vous aviez défini des moyens d'action que vous souhaitez privilégier. À l'heure de digitalisation de la société, nous souhaitons que vous puissiez consacrer un budget dédié à l'aspect numérique de la promotion de notre culture à l'étranger.

la diplomatie culturelle est un vecteur essentiel de la diplomatie d'influence. À ce titre, tous les instruments qui concourent aux politiques de coopération culturelle doivent être consolidés. hélas !, de constater que tel n'est pas le cas aujourd'hui. D'une part, les tentatives de rationalisation des moyens ont échoué. Je pense bien sûr à l'échec de l'expérimentation du rattachement du réseau culturel public à l'Institut français. D'autre part, si le contrat d'objectifs et de moyens 2017-2019 confirme l'Institut français dans son rôle d'opérateur pivot de la politique culturelle extérieure de la France, les dotations qui lui sont chaque année attribuées en loi de finances ne sont pas à la hauteur de cette ambition : nous aurons l'occasion d'en reparler très bientôt, au fil des débats budgétaires. En attendant, monsieur le secrétaire d'État, je souhaite connaître l'état de développement des outils numériques mis en place au cours des dernières années, au travers de différentes plateformes telles que Culturethèque, IFcinéma ou encore IFverso. Depuis 2013, une équipe est chargée d'approfondir ce chantier du numérique. Elle suit, en particulier, la mise en oeuvre du projet IF 360, qui donnera accès à la production culturelle française à des publics du monde entier.

Les établissements ont donc dû développer et diversifier leurs ressources en assurant des prestations de services payantes, telles que l'organisation de sessions d'examens, la location d'espaces, l'apport d'outils et d'expertise aux réseaux culturels et surtout la mise en place de cours de français.

La contrainte budgétaire imposée à l'Institut français pèse donc fortement sur les objectifs de notre politique d'influence culturelle. Or de nombreux organismes thématiques placés sous la tutelle du ministère de la culture,

Dans ces conditions, n'est-il pas envisageable de desserrer l'étau budgétaire appliqué à l'Institut français en coordonnant mieux l'intervention de tous ces acteurs ? Monsieur le secrétaire d'État, y travaillez-vous ? Dans l'affirmative, pouvez-vous nous dire quelles sont les pistes à l'étude ?

et l'Alliance française qu'a évoqué le Président de la République. Nous avons, d'un côté, l'Institut français, créé par la loi du 27 juillet 2010. Il dont la mission est de promouvoir et de diffuser la langue et la culture françaises. C'est un opérateur placé sous la tutelle conjointe du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et du ministère de la culture.

Régies par le droit local, indépendantes tant financièrement que statutairement, elles revêtent le plus souvent la forme d'associations à but non lucratif. la richesse de son action à la diversité des profils de ses antennes et à la souplesse du système associatif, tandis que l'une des forces des instituts français réside dans le pilotage de politiques culturelles. Si les instituts français et les alliances françaises sont considérés comme des réseaux complémentaires, leurs règles de fonctionnement sont donc très différentes. J'en arrive à ma question : le rapprochement concerne-t-il uniquement la Fondation Alliance française et l'Institut français à Paris,

? Dans ce cas, le rapprochement ne risque-t-il pas de brouiller la lisibilité et partant la visibilité du dispositif engagé ?

Pour les instituts français qui souhaiteraient poursuivre une mission d'enseignement en lien avec les alliances françaises, j'attire votre attention sur une synergie possible et concrète : la création d'un volontariat international d'enseignement francophone, ou VIEF. Force est de constater la disparition progressive des postes de lecteurs français à l'étranger. pénalisé notre présence, tant dans les universités locales que dans nos écoles. Il faut trouver des solutions. Ce VIEF serait une formidable occasion

Notre débat d'aujourd'hui est sans doute destiné à sanctionner sa nature chimérique. Il faut rappeler que la loi de juillet 2010 consacrait l'Institut français comme « l'opérateur pivot de l'action culturelle de la France à l'étranger » et que la loi de juillet 2016 le plaçait sous la double tutelle des ministères chargés des affaires étrangères et de la culture. Dans la pratique, les moyens réduits du second ministère cité ne lui ont jamais permis d'assurer pleinement cette tutelle. L'apport budgétaire modeste prévu par le ministère de la culture pour l'exercice 2018

La disette favorise rarement l'échange et la collaboration. Elle pousse au contraire les survivants à défendre ce qui leur reste ! Plus généralement, et en conclusion, je m'interroge sur la volonté politique de notre pays de développer et, pis

Pourtant, l'article 2 de notre Constitution énonce que la langue de la République est le français. Voilà pourquoi j'aspire à ce que tous les enfants français à l'étranger puissent apprendre à parler français. Pour y parvenir, nous pourrions créer un « chèque éducation » à l'étranger. Ce « chèque éducation », destiné à 100 % de nos jeunes compatriotes vivant à l'étranger, permettrait à tous d'accéder à un apprentissage du français

pionniers en matière de diplomatie d'influence. C'est d'ailleurs ce qui nous permet aujourd'hui de jouer un rôle important dans certaines zones du monde ; je pense en particulier au rôle que nous jouons aujourd'hui au Moyen-Orient, qui s'appuie sur ces fondements.

je vous poserai trois questions. Tout d'abord, après l'arrêt de l'expérimentation lancée avec nos implantations culturelles dans quelques pays dans la foulée de la création de l'EPIC « Institut français », en 2011, nos instituts français sont tous aujourd'hui des établissements à autonomie financière. Ce statut est en délicatesse avec les principes de la LOLF,

échéance ? Ensuite, pourquoi imposer des plafonds d'emplois aux établissements à autonomie financière, alors que la croissance autofinancée de leurs activités est le sens même de leur mission et de leur influence ? villes comme Lisbonne ou Vienne, nos instituts siégeaient dans des lieux symboliques, qui constituaient par eux-mêmes une présence, une influence et une histoire. Nous avons vendu, ou tenté de vendre, ce patrimoine. Pouvons-nous envisager une remise en cause de cette politique d'abandon ? La parole

Dans le droit fil de notre histoire, notre politique étrangère, indissociable de notre présence sur de nombreux théâtres d'actions militaires, entend être à la hauteur d'une France qui rayonne. Si la fierté peut être de mise, sachons aussi rester modestes. Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'État, d'exprimer une inquiétude, alors que nous débattons cet après-midi du rôle et de l'avenir de l'Institut français. Cet établissement public, chargé de la délicate mission de favoriser la promotion des arts et des lettres à l'étranger, pour utiliser une expression volontairement

l'institut était en quête « d'un nouveau souffle, d'une nouvelle ambition et d'une position plus claire ». Spectacle vivant, livre, cinéma, soutien à tous les savoirs et aux idées : tels sont les secteurs d'intervention de l'Institut français, aux côtés d'un réseau de 160 services de coopération, de 124 établissements à autonomie financière et de quelque 800 alliances françaises installées sur les cinq continents. cette année encore, si ce n'est pas la peau de chagrin, c'est au moins la disette. Ne vous méprenez pas : je mesure qu'il importe de réduire la dette publique. Après avoir subi une baisse de 25 % entre 2011 et 2017, au prétexte que le numérique compenserait ce recul, les crédits alloués à l'Institut français stagneront en 2018. C'est bien et court à la fois Sans sous-estimer l'importance des réseaux sociaux, il ne faut pas céder aux dangereuses illusions que peut nourrir la multiplication des clics. Monsieur le secrétaire ne pourrions-nous pas sanctuariser ces crédits, afin de réaffirmer au monde que la patrie des droits de l'homme reste fidèle à sa vocation universaliste et aux Lumières, en même temps qu'elle n'hésite pas à être au diapason de la révolution numérique ? La parole est à M. le secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous avez

celui-ci a déjà signé une vingtaine de conventions avec des régions et des grandes villes. Aujourd'hui, toutefois, faute de moyens, l'institut ne semble plus en mesure de poursuivre cette politique de conventionnement avec les collectivités territoriales. Or cette politique présentait un intéressant effet de levier, puisque, pour un euro mis sur la table par l'institut, les collectivités territoriales abondaient d'autant. Ce mode de cofinancement nous a d'ailleurs longtemps été présenté comme l'une des solutions miracles à la baisse des subventions publiques. pour que cofinancement il y ait, il faut une mise de départ minimale ! Or, aujourd'hui, faute de moyens pour l'Institut français, l'effet de levier fonctionne à l'envers pour tout euro que l'institut n'est plus capable de mettre sur la table, c'est autant de financements des collectivités territoriales qui sont perdus pour l'action culturelle extérieure. En 2014, quelque 3,12 millions d'euros avaient été mobilisés sur ce dispositif, dont 1,4 million d'euros de mise de fonds initiale de l'Institut français.

quelles actions concrètes le Gouvernement peut-il mettre en place pour renverser ce cercle devenu vicieux ? Quelles sont les perspectives de collaborations futures entre les collectivités territoriales et l'Institut français ? Excellente question ! La parole est

ce type avec l'Institut français, pour promouvoir à l'international des créateurs ou des opérateurs culturels implantés dans ces territoires

et ses créateurs, alors que notre politique dans ce domaine est, malgré tout, relativement modeste. Il est indispensable de renouer avec une politique de promotion de la francophonie, mise en retrait ces dernières années. La coopération linguistique, le soutien aux lycées français à l'étranger, notre rôle dans les institutions francophones, la place des instituts de recherche dans le monde et le développement du français sur internet, dans les médias, les livres et le cinéma doivent être renforcés, dans notre intérêt comme dans celui de nos acteurs culturels et économiques. Comme l'avait proposé le Président de la République durant sa campagne, l'Institut français pourrait évoluer vers une grande agence culturelle internationale. L'enseignement du français et en français n'est pas une valeur du passé ; c'est un vecteur essentiel de notre influence, mais aussi de la lutte contre la diffusion du radicalisme. Des moyens importants devront lui être consacrés, en particulier en Afrique.

Il ne s'agit pas d'être méprisant vis-à-vis de l'action des pères fondateurs de la francophonie, qui a été remarquable. Il s'agit de s'adapter, pour que notre jeunesse

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question porte sur le modèle économique de l'Institut français. Les moyens de l'Institut français se sont en effet considérablement réduits depuis sa création. L'État demande par ailleurs à l'institut de de diversifier ses ressources propres, issues du mécénat et de cofinancements de la Commission européenne et des collectivités territoriales. L'apport de ces ressources propres reste limité et très variable dans le temps. Elles sont passées, entre 2016 et 2017, d'environ 15 % à environ 12 du budget de l'Institut français. La concurrence est vive, et le mécénat beaucoup plus dynamique dans certaines parties du monde que dans d'autres ; enfin, il fait toujours naître le risque de créer

Le développement de cours de français en ligne est envisagé : combien cette activité est-elle susceptible de rapporter ? Enfin, les compétences de l'Institut français dans le domaine de l'expertise culturelle ne pourraient-elles pas être davantage valorisées ? La parole est à M. le

Les ressources propres ne doivent donc pas être conçues comme venant se substituer à l'argent public, mais comme venant l'accompagner et permettre d'en démultiplier l'impact.

alors que, simultanément, la demande de culture française est toujours aussi forte dans le monde. C'est à l'aune de ce double constat que nous devons décider ce que nous voulons faire de notre réseau d'opérateurs à l'étranger. de vue, ce débat sur l'avenir de l'Institut français est bienvenu. Il pose deux questions. Celle, tout d'abord, de la restructuration du réseau culturel français. Lors de son audition, le 24 octobre dernier, par notre commission, Jean-Yves Le Drian a en effet affirmé étudier « la pertinence d'un rapprochement entre l'Institut français et la Fondation Alliance française, afin de favoriser les synergies et de décupler notre action dans le domaine culturel ». Deux conventions, de 2010 et 2012, portant sur le rapprochement des identités visuelles et les synergies à rechercher avaient permis d'amorcer cette restructuration. Force est cependant de constater que, sept ans plus tard, ce rapprochement n'est pas allé très loin. La seconde question posée par le débat est celle des moyens financiers. En février dernier, Jacques Legendre et moi-même avions souligné la contradiction, au contrat d'objectifs et de moyens 2017-2019, qui pouvait exister entre la restructuration en cours et les moyens de plus en plus modestes. En effet, depuis sa création, en 2011, les crédits totaux dévolus à l'Institut français ont diminué de 25 % et ses crédits d'intervention, de 34 %. Quant au ministère de la culture et de la communication, sa dotation n'est que de 2,3 millions d'euros. De surcroît, les ressources complémentaires restent marginales pour compenser le déclin structurel des crédits alloués à l'institut. Si l'une des composantes concernées se trouve à ce point contrainte financièrement, il est à craindre que ce rapprochement ne puisse être mené dans de bonnes conditions. Monsieur le secrétaire d'État, à l'heure où la concurrence en matière d'offre linguistique s'intensifie- vous avez parlé des centres Confucius, mais il y a aussi tous nos partenaires européens, avec lesquels nous sommes malheureusement en concurrence -, comment pouvons-nous

qui porte un message universel et dont la culture rayonne dans le monde. Hélas, lorsque le déficit dérape, nos dirigeants ont une fâcheuse tendance à se servir du patrimoine immobilier national comme variable d'ajustement, y compris quand il s'agit de bâtiments emblématiques et symboliques ! La vente de trésors nationaux comme le palais Clam-Gallas de Vienne ou la maison Descartes à Amsterdam a constitué une erreur majeure, non seulement en termes de visibilité et de rayonnement pour notre pays, mais aussi en termes de stratégie, puisque la France doit désormais louer à prix d'or des bâtiments pour ses différents services et représentations. Il faut stopper l'hémorragie et il n'est pas trop tard, monsieur le secrétaire d'État ! La France saura-t-elle éviter de renouveler cette faute dans où le bâtiment qui abritait notamment l'Institut français et l'Alliance française est vide et invendu depuis plus d'un an an ? Plus largement, le Gouvernement ne pourrait-il pas envisager la création d'un groupe de réflexion composé de parlementaires, de personnalités du monde de la culture et de l'économie, qui serait chargé de repenser la gestion immobilière de l'Institut français et du réseau culturel français dans le monde ? Il ne faut pas reproduire les erreurs du passé ! Il faut chercher des solutions innovantes pour maintenir notre patrimoine à l'étranger grâce à la recherche de partenariats avec le secteur privé, le monde associatif et le monde économique. Il y va du rayonnement et de l'influence de la France ! La parole

qui nous ont permis de préserver un patrimoine monumental, je dirai même majestueux. Vous le savez, nos services culturels à New York sont hébergés dans un magnifique bâtiment, un hôtel particulier qui se trouve en face de Central Park. Grâce à l'action d'Antonin Baudry il y a quelques années,

Cantonné à une offre essentiellement artistique de la France, l'Institut français s'est malheureusement peu à peu ossifié, a vu ses moyens rognés, faute d'une lecture claire des objectifs à atteindre et malgré de très nombreuses compétences internes.

Il convient de transmettre des messages cohérents qui font écho aux positions internationales de la France. La réduction des budgets, d'une part, le changement de paradigme qu'impose l'Agenda 2030 du développement durable, la concurrence des modèles de civilisation et les enjeux économiques auxquels sont confrontés nos grands opérateurs économiques, d'autre part, obligent désormais la France à dessiner un schéma synergique. Ce schéma doit rassembler autour de l'Institut français l'ensemble de nos réseaux scolaires, universitaires, éducatifs et culturels,

dans un contexte budgétaire que nous savons contraint à l'aide publique au développement de notre pays, dans une acception large et assumée

chargé de porter une ambition renouvelée par la diplomatie d'influence contribue au rayonnement de la France à l'étranger, dans un dialogue renforcé avec les cultures étrangères, dans un souci d'écoute, de partenariat et d'ouverture. Depuis la promulgation de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine en juillet 2016, le ministère de la culture partage à nouveau la tutelle de l'Institut français avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Alors que l'Institut français est reconnu comme un outil d'influence et de coopération, mais également comme un pôle d'expertise et de conseil, je constate avec satisfaction que l'action culturelle extérieure de l'État est citée en troisième position dans la feuille de route qui vous est fixée par le Premier ministre. Pourtant, en dépit de tous ces beaux signaux très positifs, le ministère de la culture demeure un très piètre financeur de l'Institut : moins de 2 millions d'euros en 2018 pour un budget de près de 3 milliards d'euros, soit une subvention quatorze fois moins élevée que son autre ministère de tutelle Peut-être devrions-nous prendre exemple sur nos voisins allemands, qui n'hésitent pas à faire du en faisant appel à des financements extérieurs à l'État. Je crois tout de même qu'il faut prendre conscience que l'Institut français va bien au-delà des missions qui sont les siennes. Nous avons pu le constater au cours de nos déplacements

et le Centre national d'enseignement à distance. Une coordination et une mutualisation des moyens seraient facteur d'efficacité. Deuxièmement, il paraît essentiel d'élaborer des plateformes communes à tous les organismes qui concourent au rayonnement de la langue française et de la francophonie à l'étranger,

de nouvelles formes de pédagogie et d'aide à la consultation et à l'apprentissage doivent être développées. Quatrièmement, l'Institut français d'Agadir dispose d'un théâtre en plein air, seul lieu capable d'accueillir trois cents personnes, qui n'est pas couvert et qui est donc difficilement utilisable. Il est impossible à l'institut de réaliser une couverture sur ses fonds propres.

que doivent passer les étudiants étrangers dans le cadre des opérations Campus France. Certains instituts français peuvent faire passer ces tests, d'autres non. Celui d'Agadir joue un rôle opérationnel de collecte des informations d'aide à l'établissement des dossiers, mais ne peut pas procéder lui-même à la réalisation des tests, qui doivent être effectués à Marrakech. La plus grande université du Maroc, avec 150 000 étudiants,

La mission de l'Institut français est de développer l'influence et l'attractivité de la France par la promotion de sa culture et de sa langue. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 300 millions de francophones dans le monde.

Pour que le français demeure la langue de l'excellence culturelle, il faut relancer son apprentissage et renforcer sa place à l'étranger. Le Président de la République l'a rappelé : pour lui, la francophonie est essentielle et constitue un sujet majeur.

Certes, d'autres acteurs agissent également pour la promotion de la langue française à l'étranger, comme les différentes Alliances françaises, qui sont des émanations de la société civile, ou l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une institution politique, mais l'Institut français reste le seul service culturel de la France. Monsieur le secrétaire d'État, entendez-vous donner les moyens à l'Institut français de demeurer un acteur de la mise en oeuvre de la politique francophone du Président de la République ? Ne pensez-vous pas souhaitable que la Fédération internationale des professeurs de français, qui oeuvre aujourd'hui pour la promotion de notre langue dans les systèmes d'éducation locaux, soit associée à l'Institut français dans le cadre d'une coopération rapprochée et pérenne, notamment dans les pays où le français est en recul

J'ai longtemps ignoré que j'étais francophone ... « Français sans problème, « Il me faut donc vivre la francophonie en surplus « Et pour mieux dire en conscience ... « Si je perds cette conscience, « La francophonie cesse d'être en moi. Si tous les francophones la perdent, « Elle cesse absolument d'être ... « La francophonie n'a pas de papiers, « Elle n'existe que si à chaque génération « Des hommes se reconnaissent francophones

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. La commission qui a demandé ce débat disposera d'un temps de parole de dix minutes, y compris la réplique, puis le Gouvernement répondra pour une durée qui ne

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

réalisé. Nous avons cherché à répondre à plusieurs interrogations : la nouvelle géographie prioritaire est-elle pertinente ? Comment sont pris en charge les quartiers sortants ? Comment sont mis en place les contrats de ville ? Les acteurs de la politique de la ville ont-ils été au rendez-vous ? Quel est leur niveau d'engagement ? Les crédits spécifiques de la politique de la ville interviennent-ils en complément des crédits de droit commun ?

Néanmoins, nous avons constaté lors de nos déplacements que ces critères ne permettaient pas de prendre en compte certains territoires moins denses, comme le bassin minier, ou des poches de pauvreté enclavées dans des zones de mixité sociale. Nous avons recommandé au Gouvernement d'identifier les poches de pauvreté non retenues dans la géographie prioritaire en raison du seuil d'habitants et d'évaluer si elles nécessitent la mise en place d'outils spécifiques. place d'outils spécifiques. Pour les quartiers sortants, c'est-à-dire ceux qui ne répondent pas aux critères de la nouvelle géographie prioritaire, la loi Lamy a mis en place un dispositif de veille active. Or nous avons constaté que les moyens et le suivi de ces quartiers sont insuffisants. Il nous paraît important que tous les quartiers sortants fassent l'objet d'un suivi par l'État, indépendamment de l'existence d'un contrat de ville. Ce suivi permettra de savoir

J'en viens aux contrats de ville, qui mettent en oeuvre la politique de la ville. Quelque 435 contrats de ville ont été signés. Ils reposent sur trois piliers, qui permettent d'assurer une meilleure cohérence entre les actions menées au titre du volet économique et social et celles qui sont menées au titre du volet urbain. Les modalités du pilotage des contrats de ville à l'échelle intercommunale sont globalement satisfaisantes. Néanmoins, l'impact des réformes territoriales sur la mise en oeuvre de ces contrats, notamment en Île-de-France, devra faire l'objet d'un examen attentif. Au titre du pilier « cohésion sociale », nous avons choisi de porter notre attention sur la tranquillité publique, question récurrente des habitants des quartiers prioritaires. Outre que les services de police et la justice doivent amplifier leurs actions pour assurer la tranquillité des habitants dans ces quartiers, les bailleurs sociaux ont eux aussi un rôle à jouer, notamment

toutefois dans certains quartiers l'échec des politiques publiques. Les conditions de vie des habitants et celles des personnels de proximité sont devenues dangereuses et la mise en place d'une zone de sécurité prioritaire ne suffit pas toujours. Il ne faut pas abandonner ces quartiers « en difficulté extrême ». Nous proposons, au contraire, qu'ils fassent l'objet d'un traitement global des difficultés qui nécessitera un renforcement des moyens de droit commun, lequel ne peut se faire au détriment des autres quartiers. un mot du volet économique. La question de l'emploi est fondamentale dans les quartiers, où le taux de chômage est largement supérieur à la moyenne. Nous considérons qu'il ne faut pas opposer les aides à la personne aux aides en fonction de l'implantation géographique des entreprises. Autrement dit, il ne faut pas opposer emplois francs et zones franches urbaines. Une réflexion sur ces deux formes d'actions doit être menée en toute transparence, afin de retenir les dispositifs les plus efficients.

de coconstruction avec les habitants est un axe majeur de la loi Lamy, qui trouve sa traduction au travers des conseils citoyens et des maisons de projet dans le cadre du NPNRU. Le conseil citoyen a pour vocation de réunir, au sein d'une même instance, des habitants des quartiers tirés au sort et des représentants des associations, comme des acteurs locaux. Certains élus ont pu faire preuve d'une certaine réticence à le mettre en place, notamment lorsque préexistaient dans certains territoires des instances de participation ou lorsque la mise en place de précédents dispositifs participatifs avait échoué. 1 054 conseils citoyens ont été recensés et trois quartiers prioritaires sur quatre sont couverts. Néanmoins, le conseil citoyen nous a paru être encore une instance balbutiante.

la loi Lamy a prévu la mise en oeuvre d'un nouveau programme national de renouvellement urbain centré, en priorité, sur les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants. Ainsi, 216 quartiers ont été retenus. En complément, 274 quartiers dits « d'intérêt régional » ont été choisis, pour lesquels l'ANRU interviendra, mais dans une moindre mesure. S'agissant du financement du NPNRU, chacun s'accorde à dire que l'enveloppe de 6 milliards d'euros était insuffisante. Les acteurs locaux nous ont fait part de leurs doutes sur l'ambition de ce programme et ont partagé leur crainte de voir leur projet contraint. Comment, dans ces conditions, mobiliser les habitants pour coconstruire le projet ? Nous avons proposé, avec Valérie Létard, de porter le montant du NPNRU à 10 milliards d'euros et de rétablir la parité de financement entre l'État et Action Logement. Nous avons été partiellement entendues, puisque le projet de loi de finances prévoit que le montant du NPNRU soit porté à 10 milliards d'euros, dont un milliard d'euros, monsieur le ministre, sera financé par l'État. Toutefois, les modalités de financement de ces 4 milliards d'euros supplémentaires ne sont pas actées à ce stade. S'il semble acquis, en effet, qu'Action logement participera à hauteur de 2 milliards d'euros supplémentaires, la participation des bailleurs sociaux est, pour l'heure, incertaine en raison des débats sur la réforme des aides personnalisées

Afin d'éviter une déperdition de concours financiers, nous souhaitons également rendre possible, pour ces quartiers d'intérêt régional, l'insertion, dans les conventions ANRU-région, d'une clause de revoyure qui permettrait, à mi-parcours, de redéployer des crédits au sein d'une région.

rénovation du NPNRU, qui s'inscrivent dans la continuité du PNRU, le réexamen du dispositif de, qui pénalise les communes les plus vertueuses, ainsi que le réexamen des montants des aides octroyées aux bailleurs sociaux. Nous espérons que l'augmentation du montant du NPNRU permettra ces assouplissements et que sera privilégié le recours aux subventions plutôt qu'à des prêts bonifiés, sous peine d'accroître plus encore l'endettement des communes.

Pour favoriser cette mixité sociale, nous pouvons agir sur les attributions de logements sociaux, en veillant à ce que les ménages les plus modestes ne soient pas systématiquement orientés vers les quartiers faisant l'objet d'un programme de rénovation urbaine. À ce sujet, je dois vous l'avouer, nous craignons que, dans le cadre du projet « Un

». Nous croyons qu'il faut aussi prendre en compte cette situation. Quant au traitement des copropriétés, il constitue l'un des défis majeurs du NPNRU. Nous souhaitons qu'il soit remédié à l'absence de recensement exhaustif des copropriétés situées dans En outre, nous estimons que des outils mieux adaptés doivent également être mis en place pour faire face à l'augmentation du nombre de copropriétés en difficulté. En conclusion, monsieur le ministre, nous avons estimé que si la réforme de la politique de la ville était bien engagée, elle souffrait cependant d'un manque de

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs,

pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le Président de la République est intervenu, le 14 novembre dernier, dans la métropole européenne de Lille, pour fixer le cap d'une politique de la ville renouvelée. Depuis quarante ans, tous les gouvernements se sont évertués à trouver des solutions, afin de gommer les inégalités entre la périphérie et le centre de nos métropoles. Pourtant, aujourd'hui encore, plus de 5 millions de nos concitoyens vivent dans des quartiers dits « de géographie prioritaire », dont le revenu moyen par habitant est inférieur de 60 % au revenu médian, c'est-à-dire à 11 250 euros par an. Les collectivités locales et leurs élus sont en première ligne du combat quotidien pour faire en sorte que ces territoires, et surtout leurs habitants, ne décrochent pas totalement. Je m'appuierai sur le cas de la métropole européenne de Lille pour illustrer le travail des pouvoirs publics locaux. La métropole européenne de Lille pilote l'un des plus importants contrats de ville français. Il concerne 360 000 habitants. Ce contrat de ville inclut un programme de renouvellement urbain à dix ans. Dans ce cadre, 7 000 logements devraient être traités, qu'ils soient détruits, reconstruits ou réhabilités. Des incertitudes pèsent sur ce programme, dont les deux tiers dépendent des capacités d'autofinancement ou d'emprunt des bailleurs, notamment à cause d'un manque de visibilité. Monsieur le ministre, ma question porte sur les modalités de mise en oeuvre des annonces du Président de la République et sur la place qui sera faite aux collectivités locales. Sur la forme, dans la définition du plan de bataille voulu par le Président de la République et pour lequel il a confié une mission à M. Jean-Louis Borloo, quelle place sera faite aux collectivités locales et, en premier lieu, aux intercommunalités, qui sont les pilotes de ces contrats de ville ?

M. le ministre. Monsieur le sénateur, vous m'avez interrogé sur la place qui sera faite aux collectivités locales dans ce dossier particulièrement important. On ne peut agir sur la politique de la ville

De plus, les collectivités locales, quelles que soient les strates, ont un impact important et indispensable sur la politique de rénovation de ces quartiers.

a décidé de mettre en place un conseil présidentiel de la ville. Il fait ainsi la démonstration d'une volonté très forte de faire de ce dossier un enjeu national. Ce conseil devrait se réunir à l'Élysée tous les trois mois.

Aux termes de la loi de programmation de 2014, le QPV correspond à un espace urbain continu regroupant au moins 1 000 habitants et dont le revenu médian est défini comme critère unique de classification. Or la référence à ce revenu médian apparaît aujourd'hui pénalisante pour des communes avec des quartiers très défavorisés et les fait sortir de la classification QPV issue de la nouvelle géographie. En effet, d'une certaine manière, des méthodes de calcul du revenu moyen médian

Or le territoire de l'ex-bassin minier du Nord-Pas-de-Calais se caractérise par un habitat spécifique en « cités », nettement moins dense que les barres HLM, et par une pauvreté diffuse : l'écart entre les revenus est donc moins important que dans d'autres territoires entre ces quartiers et le reste de la ville. Vous admettrez que cette double peine est difficile à admettre pour les élus locaux L'approche antérieure à 2014, fondée sur des critères multiples- minima sociaux, taux de familles monoparentales, taux de chômage, pourcentage de la population sans diplômes ... -était donc plus juste, parce que plus proche de la réalité. Je souhaite donc savoir, monsieur le ministre, si vous entendez intervenir auprès des services de Bercy afin de faire évoluer les critères de classification. Dans la négative, envisagez-vous des mécanismes correctifs ? J'ajoute, pour conclure, que cet infléchissement de la législation serait en cohérence avec les engagements pris par l'État dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais signé en mars dernier par le Premier ministre, M. Bernard Cazeneuve. est à M. le ministre. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur des critères qui ont été définis par la loi de 2014. Dans ce texte, il est mentionné qu'il n'est pas prévu d'actualisation de la géographie prioritaire avant 2020, ce qui correspondra à l'achèvement de la nouvelle génération des contrats de ville, afin que ceux-ci puissent produire tous leurs effets. que cette définition de la géographie prioritaire sur la base d'un critère unique permet tout de même de faciliter son actualisation.

sinon vous rassurer, du moins vous dire que nous sommes très attentifs à ce qui se passe sur votre territoire. Vous avez rappelé le contrat concernant le bassin minier signé par le Premier ministre Bernard Cazeneuve au mois de mars 2017. J'ai eu

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 48 millions d'euros, tel est le montant investi par l'État pendant les dix dernières années sur la politique de la ville. 48 millions d'euros pour retrouver, même s'il y a eu des réussites qu'il ne faut pas nier, des quartiers où règne la violence au quotidien, où la désespérance est généralisée, où le chômage est endémique.

à faire preuve de concision dans la rédaction législative. Plus sérieusement, je conviens qu'il y a une grande complexité de nos procédures. Je vous entends

son souhait de voir rouvrir les internats d'excellence dans les zones rurales et dans les quartiers difficiles. Lancés en 2000 dans le cadre du plan de relance de l'internat scolaire public, puis promus à la suite de la dynamique Espoir banlieues de 2008, ils ont rencontré un fort succès et le bilan est très largement positif au regard de l'amélioration des résultats scolaires des adolescents internes. Toutefois, jugés trop couteux par la précédente majorité, les internats d'excellence ont été dissous dans les autres internats, plus précisément dans le dispositif des internats de la réussite.

action sociale auprès des habitants et action urbaine -, qui constitue les deux pieds de cette politique depuis sa création. Or, cet été, que Philippe Rio, initiateur de l'appel de Grigny, qualifie d'« été meurtrier », vous avez procédé à une triple attaque des fondements de cette politique.

Combien d'associations n'ont pas pu assurer leur rentrée ? Avez-vous un chiffre à nous communiquer, monsieur le ministre ? Il serait intéressant d'en débattre. Nous ne pouvons accepter cette décision d'autant plus que vous avez opéré- c'est le deuxième volet de cette attaque -une suppression de crédits, à hauteur de 46,5 millions d'euros. Là encore, combien de projets utiles ont été stoppés en raison de cette nouvelle coupe, qui se conjugue avec la baisse des dotations aux collectivités territoriales ? Enfin, en attaquant la prétendue rente des offices d'HLM, ce gouvernement pénalise directement la construction et la réhabilitation des immeubles dans ces quartiers, puisque les bailleurs sont les principaux financeurs de la rénovation urbaine.

quand allez-vous arrêter de nous annoncer des milliards d'euros qui n'existent pas ? Pensez-vous concrètement pouvoir aller plus loin pour l'ANRU que le simple engagement des 15 millions d'euros prévus

La parole est à M. Daniel Dubois, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour réellement changer nos quartiers prioritaires,

Il faut donc assurer dès le départ une nouvelle mixité, à travers une politique de peuplement adaptée. C'est très difficile à faire.

Toutes ces actions doivent être menées de façon concomitante. Dans ces quartiers, les politiques publiques d'accompagnement de proximité sont essentielles et doivent être contractualisées entre tous les acteurs

le devoir des familles pour assurer la parentalité : c'est un enjeu majeur mais particulièrement difficile, compte tenu de ce que nous savons sur les renouvellements de population dans un certain nombre de ces quartiers.

le plus efficace de la politique déconcentrée de l'État dans ces quartiers. Pour les avoir presque tous rencontrés en les réunissant

quartiers. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quand nous légiférons pour les 5 millions d'habitants des quartiers populaires, nous devons avoir à l'esprit l'ampleur des inégalités qu'ils subissent un taux de pauvreté à 42 %, un taux de chômage à 27 %, souvent des logements insalubres. Ces inégalités sociales ont un impact direct sur l'état de santé des habitants : l'espérance de vie à la naissance y est, par exemple, beaucoup plus faible. Face à cette urgence sociale, notre responsabilité collective est engagée. Il est de notre devoir de tenir la promesse républicaine d'égalité sur notre territoire. Nous le devons aux habitants. C'est un principe de justice sociale ; c'est aussi une question de dignité. Vous le savez, les habitants de nos quartiers populaires ne sont pas des oisillons qui attendent la béquée. Ce sont des citoyens qui souhaitent simplement qu'on leur offre les mêmes chances de réussite. Quand, le 13 novembre dernier à Clichy-sous-Bois ou le 14 à Tourcoing, j'ai écouté le Président de la République et pris connaissance des mesures qu'il proposait pour les 5 millions d'habitants de nos quartiers, pour eux, j'ai eu envie d'y croire

de la faiblesse des financements qui rendent tout engagement inatteignable ou insincère. En ces temps où la parole politique est dévalorisée, c'est jouer avec le feu que de ne pas respecter ses engagements. Veillez à ne pas en rester au stade des incantations et des effets d'annonce. Monsieur le ministre, le 24 octobre dernier, vous avez confirmé l'engagement de l'État, décidé par le précédent gouvernement, dont Patrick Kanner faisait notamment partie, de 1 milliard d'euros pour la rénovation, indiquant ainsi votre engagement annuel de 65 millions d'euros. Comment expliquer alors que, pour 2018, nous ne soyons qu'à 15 millions d'euros ? Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer une estimation du nombre d'emplois francs qui seront signés en 2018 ? La parole

tout à fait normal que nous travaillions tous à cet objectif, mais il est difficile à atteindre compte tenu de la situation que nous avons constatée. Nous allons faire le maximum pour aller dans ce sens. Vous avez une crainte sur les finances

! C'est moi qui préside la séance, mon cher collègue, et j'allais dire que M. le ministre avait quasiment épuisé son temps. La parole est à Mme Michèle Vullien, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dès que l'on évoque la politique de la ville apparaît une problématique qui me tient tout particulièrement à coeur et qui concerne les enjeux de mobilité. Nous savons que Mme Élisabeth Borne organise en ce moment les Assises de la mobilité partout en France. Sans vouloir interférer dans ses travaux, il est nécessaire de réaffirmer l'impérieuse nécessité d'offrir des solutions de déplacement et de transport aux populations les plus modestes ou aux territoires les plus enclavés, pour ne pas dire. La réponse à ce besoin passe nécessairement par un portage politique volontariste de sortir du « tout-voiture », répondant par la même occasion à des contraintes environnementales désormais prioritaires, et par la capacité de nos différentes strates administratives compétentes de renouer le dialogue, loin des clivages politiques partisans, uniquement porté par l'intérêt général.

sous toutes leurs formes, font partie intégrante des solutions d'avenir pour notre planète et que l'équité territoriale doit engendrer, demain, une ville sans couture ? La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi de 2014 a fait rentrer dans la politique de la ville, grâce au critère unique du revenu par habitant, des quartiers situés en zones rurales. Patrick Kanner a mis en oeuvre avec efficacité cette politique, je peux en témoigner à Auch. Le Président de la République a indiqué vouloir mieux cibler l'action de la politique de la ville sur les quartiers en très grande difficulté. Si cette décision se comprend au regard des principes et valeurs de la République qui nous rassemblent, pouvez-vous nous rassurer, monsieur le ministre, sur le maintien dans le dispositif, de façon durable dans le temps, des quartiers politique de la ville situés en zones rurales ? Il est en effet essentiel que l'action collectivement déjà engagée, qui a souvent déjà produit des effets positifs et qui suscite légitimement de fortes attentes des citoyens, des associations et des élus, ne soit pas déçue. finances pour 2018 de 15 millions d'euros de crédits de paiement pour l'ANRU laisse comprendre que très peu de projets de renouvellement urbain seront réalisés et financés en 2018. Est-ce à dire que l'année 2018 sera consacrée au mieux à des études, au pire à rien ? S'il en est ainsi, quel message faites-vous passer aux habitants de ces quartiers ? Comment l'État, par le truchement de l'ANRU, va-t-il compenser le désengagement ou l'affaiblissement de nombreux acteurs comme les bailleurs sociaux, les départements et les régions ? Le calcul de la participation de l'ANRU au financement va-t-il être revu à la hausse pour opérer les nécessaires compensations ? Enfin, dans une perspective d'aménagement du territoire moderne, le temps n'est-il pas venu de penser différemment les stratégies d'accueil et de peuplement à partir d'une relation « métropole-territoires ruraux ou périphériques » qui permettrait de donner un sens concret au principe d'égalité des territoires auquel nous sommes tous attachés ? La parole est à M. le ministre.

Le Gouvernement n'entend pas modifier la liste des quartiers qui ont été retenus dans le cadre de la

territoires ruraux. Je sais, pour avoir signé un contrat dans le Gers en présence de la métropole et et du pays présidé par votre collègue Raymond Vall, que vous êtes très allant dans ce domaine. Nous ne pouvons qu'inciter toutes les métropoles, métropoles, y compris les plus célèbres, à pratiquer une politique du ruissellement qui favorisera tous les territoires ruraux. La parole est à M. Joël Labbé, pour le groupe du Rassemblement

ne doit pas être vue comme un obstacle et une source de délais supplémentaires, mais comme une possibilité d'améliorer le projet comme d'éviter des risques de blocages ou d'insatisfaction ultérieurs. Nous multiplions régulièrement les instances de consultation et de participation des citoyens. Nous en avons d'ailleurs inscrit le principe dans notre Constitution, l'article 7 de la Charte de l'environnement. Nous l'avons confirmé en ratifiant plusieurs traités internationaux. Cette participation se pratique aujourd'hui dans des domaines diversifiés, en particulier l'environnement et l'urbanisme. Le dispositif des conseils citoyens a été qualifié d'« instance balbutiante » par les auteurs de ce rapport ma question est simple : comment envisagez-vous de renforcer les conseils citoyens, de les conforter dans leur mission et d'engager une mise en cohérence des différents systèmes de participation des habitants sur les territoires ? La parole est à M. le ministre.

les difficultés pratiques de renouvellement. Il faut aujourd'hui tirer le bilan du fonctionnement des conseils citoyens. Pour avoir rencontré depuis quatre

à restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants. À l'occasion des quarante ans de la politique de la ville, le 6 octobre dernier, le Gouvernement a souhaité donner un nouvel élan à la politique de la ville et s'est engagé à augmenter de 1 milliard

En parallèle, l'article 52 du projet de loi de finances pour 2018 impose, en contrepartie de la baisse des APL de 60 euros dans le logement social, une réduction des loyers de solidarité, qui sera finalement étalée sur trois ans. Pour l'année 2018, la baisse des loyers correspondra toutefois à une perte de 822 millions d'euros. Cette perte devra être absorbée par les offices publics de l'habitat, qui détiennent 2,5 millions de logements. Cette mesure, qui intervient en pleine négociation du futur NPNRU pour les années 2018-2024, a des effets directs sur la capacité d'autofinancement des organismes d'HLM et va nécessairement fragiliser la politique locale en faveur du logement social. Je m'inquiète donc de la capacité des bailleurs à investir au cours des prochaines années dans les quartiers prioritaires et des incidences de ces mesures sur la réalisation des projets engagés dans le cadre du NPNRU. Pouvez-vous, monsieur le ministre, me préciser aujourd'hui les contreparties qui seront données aux bailleurs sociaux afin de limiter l'impact de ces mesures sur l'ensemble de la chaîne de production de logements ? Les engagements de l'État en matière de rénovation urbaine pourront-ils être tenus ? La parole est à M. le ministre.

Vous avez évoqué les contreparties. Nous sommes justement en train de finaliser un certain nombre de propositions qui me permettent, là aussi, de vous adresser un message rassurant.

la perte pour les six bailleurs sociaux qui suivent le projet ANRU est de 21 millions d'euros par an. Je ne suis donc pas certain que les engagements qui ont été pris lors du protocole de préfiguration

parmi les dix objectifs de la politique de la ville fixés par l'Observatoire national de la politique de la ville figure en sixième position : « Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance. devenus des zones de non-droit dans lesquelles la tranquillité des habitants est contrariée, pour ne pas dire mise à mal, par nombre d'actes délictueux et des commerces illicites. Le trafic de stupéfiants en est certainement l'illustration la plus parlante, une réelle économie parallèle s'installant même dans ces quartiers.

avoir proposé des parcours de vie et d'insertion et à nous être entendus répondre que leur activité était sans doute beaucoup plus lucrative que tel ou tel parcours ? Dans les cellules de veille auxquelles nous participons, nous mesurons que le droit à la tranquillité et à la sécurité n'est pas forcément le même pour tous. Le Président de la République a insisté sur ce sujet lors de son déplacement dans la métropole lilloise le 14 novembre dernier, en évoquant le lancement d'une expérimentation de la police de sécurité du quotidien dans ces quartiers dès 2018. Cette présence policière est fortement attendue par nos concitoyens et par les élus locaux. Ce déploiement se fera dans le cadre d'une stratégie de sécurité partagée par les élus locaux et par les associations, stratégie qui repose à la fois sur la prévention et la répression. Dans le Nord, et plus particulièrement dans la métropole lilloise, l'appétence est grande pour expérimenter ce dispositif et des demandes ont été faites dans ce sens. Monsieur le ministre, pour répondre aux attentes et aux interrogations des élus locaux, pouvez-vous nous préciser les contours des missions qui seront dévolues à cette police dans les QPV, les moyens spécifiques leur seront dédiés et la date à laquelle les sites retenus seront

s'agissant du renouvellement de population. Nous sommes au coeur du sujet. Vous l'avez rappelé, le Président de la République a indiqué que la politique de sécurité du quotidien serait fléchée prioritairement sur un certain nombre de quartiers fragiles que nous connaissons tous et dans lesquels nous commencerons l'action dès l'année 2018. La concertation est en cours sous l'égide du ministre d'État,

M. le ministre. Monsieur le sénateur, j'aurais été étonné que vous trouviez dans les dispositions préconisées par le Président de la République un quelconque point

j'attire votre attention, monsieur le ministre, sur les questions qui ne manqueront pas de se poser en lien avec ce qui se passe sur le budget du logement. Je sais votre investissement sur cette question et le travail que le Sénat est en train de mener, mais, attention, la vente de patrimoine et toutes ces questions risquent de poser des problèmes en termes de mixité dans ces quartiers.

Nous avons dit très clairement que nous serions au rendez-vous des besoins du NPNRU et je maintiens que cet engagement sera tenu.

Lors de la nouvelle définition des quartiers relevant de la politique de la ville, un certain nombre de quartiers ont été sortis du zonage prioritaire : l'article 13 de la loi a prévu de consolider la situation de ces territoires par la mise en place d'un dispositif de veille active. Certains de ces quartiers ont été inclus dans des contrats de ville, mais pas tous. Par ailleurs, certains autres contrats de ville ont identifié de nouveaux quartiers qui n'étaient pas intégrés, mais dont la situation sociale ou économique paraissait malheureusement suffisamment dégradée pour justifier une veille active d'un autre type afin qu'ils ne deviennent pas de futurs quartiers prioritaires.

dans nos intentions de revenir fortement sur ce dispositif, si c'est la question que vous me posiez. Favoriser l'emploi des habitants de ces quartiers dans le cadre des dispositifs existants ou que nous allons mettre en place est bien sûr une priorité.

Je vous remercie au service de la solidarité et du renouvellement urbain. Pour lutter contre les ghettos, l'enfermement, il est nécessaire d'avoir un rythme de construction de logements sociaux partout dans notre pays. La loi SRU sert à cela. Il y a deux semaines, le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat, M. Thierry Repentin, vous a remis un rapport extrêmement intéressant sur l'application de la loi SRU. Si, dans son rapport, le délégué interministériel encourage à poursuivre le travail engagé avec succès lors du précédent quinquennat, il émet aussi plusieurs recommandations.

Parmi les communes pouvant être sanctionnées, les préfets ont proposé de n'en carencer cette fois-ci que 36 % sur la période 2014-2016, alors que la proportion était de 56 sur 2011-2013, seul bilan réalisé pendant le quinquennat précédent. Le constat est le même s'agissant de l'utilisation des moyens mis à disposition des préfets : la commission est contrainte de constater que le niveau

écrit à ces mêmes préfets afin que leur action puisse être développée. Nous souhaitons être rassurés sur cette volonté politique qui va dans le sens de la solidarité territoriale.

sur les dispositions de la loi SRU en ce qui concerne ce dossier. Je demande très clairement aux préfets d'appliquer les dispositions légales et les recommandations,

matière. La parole est à M. Jean-François Husson, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, monsieur le ministre, à la mi-juillet, le rapport de nos collègues Mmes Guillemot et Létard sur l'application de la loi Lamy concluait que la réforme de la politique de la ville était « bien engagée, mais fragilisée par un manque de moyens Quelques jours après, par un décret, l'État annulait plus de 46 millions d'euros de crédits de paiement et plus de 130 millions d'euros d'autorisations d'engagement affectés à la politique de la ville, notamment sur le programme 147, c'est-à-dire des crédits destinés aux programmes d'actions des associations intervenant dans le cadre des contrats de ville. Le gel des crédits à l'échelle de mon département, la Meurthe-et-Moselle, représente 200 000 euros. Au démarrage du contrat de ville, l'État finançait avec la métropole du Grand Nancy 850 000 euros, à parité. Aujourd'hui, l'État a diminué sa participation de 200 000 euros, mais pas la collectivité. Les associations, forces vives de la politique de la ville, se voient donc pénalisées par des coupes budgétaires dans leurs subventions, parfois en raison des baisses de dotations de l'État et par la suppression des emplois aidés. des emplois aidés. Monsieur le ministre, sur la base factuelle et objective de ce constat, quelles solutions comptez-vous apporter et mettre en oeuvre pour permettre aux associations, dans le cadre des relations contractuelles nouées localement avec l'assentiment de l'État, de poursuivre leurs missions au service de la politique de la ville ?

Ce qui est important, c'est que nous avons pris l'engagement qu'il n'y en aurait plus sur les budgets suivants. Si nous avons été amenés à prendre ces décisions

Monsieur le ministre, vous avez évoqué le « coup de rabot ». Comme vous l'avez également laissé entendre, les politiques de la ville ont besoin d'un vrai coup de pouce.

Cohésion, solidarité, présence et proximité pour agir au quotidien : là, vous actionnez le bénévolat plutôt que la mise en oeuvre de moyens financiers de la puissance publique. La parole

un message imprimé en plusieurs exemplaires, signé « La Direction ». Destiné « À tous les habitants de la tour et du quartier des Izards », ce message avait pour but de les « prévenir Si vous avez- je cite -la moindre complicité avec la police qui pourra empêcher nos activités qui se passent dans le hall, vous en assumerez les conséquences. Refusez le moindre coup de main de la police ». Est-il nécessaire de préciser que le véritable auteur de ce message n'était pas la direction de Toulouse Métropole Habitat, mais bel et bien des dealers qui ont fait de ces deux immeubles le siège de leur fonds de commerce et font vivre un véritable enfer à leurs habitants. Dans leur excellent rapport, nos collègues Valérie Létard et Annie Guillemot rappellent que la question de la tranquillité publique est une demande récurrente des habitants des quartiers prioritaires. Elles proposent de renforcer la présence des gardiens et des dispositifs de médiation, chose faite en l'occurrence, mais qui se révèle parfois insuffisante. C'est la raison pour laquelle les deux rapporteurs recommandent « dans les cas les plus extrêmes, où les conditions de vie des habitants et celles des personnes de proximité sont devenues dangereuses, la mise en place d'un traitement global des difficultés Monsieur le ministre, le Gouvernement envisage-t-il reprendre à son compte cette sixième recommandation du rapport ? Si oui, pouvez-vous nous détailler les mesures concrètes qui en découleront, ainsi que les moyens humains et financiers que vous comptez leur consacrer ?

M. le ministre. Monsieur Daubresse, je ne vais pas terminer par la polémique alors que je sais que nous avons la capacité de travailler ensemble de manière très constructive.

de préparer une mission confiée à Jean-Louis Borloo, vous l'avez rappelé, et je le fais en toute confiance et avec plaisir, pour que d'ici à deux ou trois mois nous puissions,